promettait dans son programme : « Nous ouvrirons les droits à l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent. Ce droit ne sera utilisable qu'une fois tous les cinq ans. » Cette promesse a été largement amoindrie par l'ajout de conditions drastiques à l'accès à une indemnisation. Désormais, le salarié démissionnaire devra, en plus des cinq ans d'ancienneté, solliciter un accompagnement au titre du conseil en évolution professionnelle, obtenir l'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel par la commission paritaire régionale interprofessionnelle. En outre, il faudra que cette aide conserve un caractère subsidiaire par rapport aux autres dispositifs. Par conséquent, cette promesse électorale, présentée partout comme une formidable avancée, ne constitue en réalité qu'une régression. En effet, alors que Pôle emploi indemnise déjà entre 70 000 et 80 000 démissionnaires par an, selon les prévisions, seules 29 300 personnes seront potentiellement concernées par ce dispositif. En matière de communication politique, c'est assez fort, mais, vis-à-vis des salariés qui subissent le mal-être au quotidien et restent dans leur entreprise

irritabilité pour plus d'une personne interrogée sur deux. Selon lui, la moitié des Français affirment que leur emploi a un impact négatif sur leur vie familiale et sentimentale et 39 %, sur leur vie sociale. Il est bien évident que que nous sommes, pour notre part, à la recherche d'un emploi épanouissant. Le mal-être au travail est une réalité concrète et notre système de sécurité sociale, que vous souhaitez faire disparaître de la Constitution, est là pour répondre aux nouveaux besoins de la vie des salariés. Les salariés démissionnaires et les travailleurs indépendants doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les autres demandeurs d'emploi. Pour financer ces indemnisations nouvelles, les syndicats ont des propositions : Force Ouvrière suggère d'instaurer une cotisation sur les indépendants, la CGT promeut un système forfaitaire

nous devions avoir un nouveau dispositif qui aurait un caractère universel et qui aurait embrassé toutes les catégories de population et catégories de profession, pour que chacun puisse bénéficier d'une indemnité compensatrice de revenus, dès lors qu'il aurait connu

deux. Plutôt que d'augmenter le nombre de bénéficiaires par l'intermédiaire de l'extension de l'assurance chômage, il eût mieux sans doute valu étendre les bénéficiaires, soit du CIF, soit du CPF de transition, après que l'on en aurait amélioré le contenu.

de loi, 50 % de plus de personnes auront la possibilité de démissionner pour un projet professionnel de création d'entreprise ou de reconversion. Ce dispositif répond donc bien à la philosophie de ce qui a été promis pendant la campagne présidentielle. J'ajoute qu'il s'agit d'une estimation, puisque c'est une logique

M. Martin Lévrier. La commission des affaires sociales a adopté un amendement tendant à préciser que seuls les salariés ayant cotisé au moins sept ans au régime d'assurance chômage pourront bénéficier de la nouvelle allocation ouverte aux démissionnaires. Non seulement la durée de sept ans paraît trop restrictive pour ce dispositif, mais il semble préférable de ne pas inscrire dans la loi le cadre précis d'antériorité.

la rédaction actuelle prévoit des conditions, mais celles-ci paraissent encore trop faibles pour limiter les risques d'un déséquilibre financier de l'UNEDIC. En effet, l'extension de l'assurance chômage aux démissionnaires conduirait à une dépense supplémentaire de 300 millions d'euros par an. Par ailleurs, l'objectif est bien d'indemniser les démissionnaires ayant un projet de reconversion nécessitant une formation qualifiante, qui ne peut être réalisée dans le cadre de leur emploi et en mobilisant les autres dispositifs existants. Or le texte laisse supposer que le démissionnaire peut être indemnisé pour tout type de formation suivie dans le cadre d'un projet professionnel. Afin d'éviter toute dérive, il convient de préciser que la formation doit être qualifiante ou que le salarié démissionnaire suit une formation complémentaire à la suite d'une parole est à M. Martin Lévrier. Cet amendement vise à inclure dans le champ des personnes susceptibles de bénéficier de l'allocation d'assurance chômage les démissionnaires souhaitant s'établir à l'étranger en vue d'y réaliser un projet de reconversion professionnelle ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Nous souhaitons permettre à ces personnes de percevoir un revenu de remplacement pendant la période de formation précédant leur départ à l'étranger. Une fois à l'étranger, les démissionnaires cesseront de percevoir l'allocation d'assurance chômage, à l'exception de ceux qui se seront installés dans un État de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse. Il convient en effet de rappeler que l'article 64 du règlement européen du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale permet aux chômeurs qui se rendent dans un autre État européen pour y chercher un emploi de conserver le droit aux prestations de chômage pendant une durée de trois mois, laquelle peut être étendue jusqu'à six mois Le dispositif prévu par notre amendement ne vise absolument pas à encourager un prétendu « exil des forces vives ». Il s'agit de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de se lancer plus facilement dans l'aventure de l'expatriation professionnelle. Cette dernière présente de nombreux avantages : elle permet notamment d'acquérir de nouvelles compétences susceptibles de répondre aux enjeux d'une économie concurrentielle et mondialisée. Par ailleurs, il importe de souligner que les entreprises créées à l'étranger par des Français constituent un véritable atout économique pour notre pays. D'après le Conseil économique, social et environnemental, l'activité de chaque créateur d'entreprise établi à l'étranger entraînerait, en moyenne, dix-neuf emplois en France. Elle est également à l'origine de flux financiers professionnels vers notre pays. De plus, ces entrepreneurs ont recours aux produits et technologies français. Quel est l'avis de la commission ? L'objet de l'amendement

d'un CPF de transition soient en priorité des démissionnaires dont le niveau de qualification est le plus bas,

l'amendement n° 219. « Nous ouvrirons les droits à l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent. » Voilà la phrase exacte du candidat Emmanuel Macron, lors de la campagne présidentielle.

Toutefois, il n'est malheureusement pas rare que ces pratiques se fassent déjà et, dans ce cadre, l'ouverture des droits au chômage des démissionnaires est plutôt une sécurité financière qu'autre chose, même si elle constitue un transfert de responsabilité financière de l'entreprise à l'État. Ensuite, cette mesure d'ouverture pourrait constituer une solution au mal-être au travail. En effet, en l'état actuel, de trop nombreux salariés restent à leur poste au mépris de leur santé pour la simple et bonne raison qu'ils ne pourraient pas supporter financièrement le poids d'une démission sans indemnité de départ et sans allocation chômage. Dans un temps où la recherche d'emploi est particulièrement difficile et chronophage, on peut comprendre que ces salariés n'osent pas ou ne puissent pas franchir le pas. Il est essentiel de revenir sur quelques données relatives au mal-être au travail. Comme le montrait une enquête de 2011, l'absentéisme et le micro-abstentéisme sont symptomatiques d'un mal-être profond profond au travail et de dysfonctionnements au sein d'une entreprise. Ainsi, plus de la moitié des salariés avouaient avoir déjà pris un repos forcé de courte durée pour évacuer le stress, ce qui représentait 3 500 euros par salarié et par an. Une seconde étude montrait qu'un quart des salariés était en situation d'hyperstress- cela pouvait concerner plus de 40 % d'entre eux dans certains secteurs -et que la moitié des travailleurs étaient touchés par un niveau élevé d'anxiété au travail. Le mal-être au travail coûterait chaque année aux entreprises 12 600 euros. Enfin, on touche ici même au principe de ce que sont les droits au chômage. En refusant aux salariés démissionnaires l'accès aux allocations chômage, on les prive d'un droit pour lequel ils ont cotisé selon le principe du salaire différé. Au final, la montagne a accouché d'une souris. En limitant les droits des démissionnaires aux seuls salariés ayant un projet arrêté, seuls 14 000 à 23 seuls 14 000 à 23 000 sur 1 million de salariés démissionnant chaque année pourraient bénéficier du dispositif, soit 2,3 % des effectifs. Ce calcul réalisé par les organisations syndicales et patronales lors de l'accord consacré à l'assurance chômage le 22 février dernier montre clairement l'insuffisance du dispositif

met en oeuvre une promesse importante du candidat devenu Président de la République : l'ouverture aux indépendants du droit à un revenu de remplacement. C'est une avancée qui correspond à l'évolution des métiers, à l'évolution de la structure de l'économie. Cependant, cette évolution doit être accompagnée pour ne pas pénaliser ceux qui, par choix ou non, sont travailleurs travailleurs indépendants. Cet amendement vise donc à s'assurer que le décret en Conseil d'État qui fixera les mesures d'application comme les conditions de ressources et de durée antérieure d'activité prenne en compte la diversité des métiers. Peut-on traiter de la même manière un indépendant agricole, dont le revenu est,

M. Martin Lévrier. Pour actualiser le mode de financement de l'assurance chômage, c'est-à-dire faire correspondre ce mode de financement à l'économie d'aujourd'hui, mais aussi à la diversité des revenus, le Gouvernement prévoit de supprimer les cotisations d'assurance chômage et de les remplacer de manière pérenne par une fraction d'une imposition de toute nature. La commission des affaires sociales a adopté à l'article 30 un amendement maintenant ouvertes plusieurs pistes de financement de l'assurance chômage, y compris les cotisations salariales. Ce choix entre en contradiction avec l'alinéa 13 de l'article 28. notre groupe propose un amendement de coordination avec l'article 30, visant à supprimer la mention selon laquelle l'allocation des travailleurs indépendants sera financée exclusivement par les impositions de toutes natures affectées à l'UNEDIC.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car cette mention est superfétatoire. Les dépenses afférentes à l'allocation des travailleurs indépendants, l'ATI, représenteront moins de 0,5 % des dépenses du régime d'assurance chômage alors que les impositions de toutes natures affectées à l'UNEDIC représenteront représenteront plus d'un tiers des ressources du régime, soit environ 13 milliards d'euros par an. Il n'est donc pas utile de préciser que le financement de l'ATI se fera exclusivement par ces impositions de toutes natures. Elles seront nécessairement couvertes par les impositions de toutes natures.

Tourenne. Il s'agit de trouver un moyen de lutter contre la multiplication des contrats précaires, lesquels ont augmenté de 165 % entre 2000 et aujourd'hui.

parole est à M. Martin Lévrier. Pour améliorer notre système d'assurance chômage, nous devons avoir deux priorités : lutter contre les emplois instables, d'une part ; faire payer les entreprises qui font supporter un coût anormal au système, d'autre part. cela est indiqué dans une note du Conseil d'analyse économique, les contrats courts sont fréquemment des réembauches par un ancien employeur. Ce fut le cas de plus de 70 % des réembauches en CDD en 2011. Les entreprises qui n'offrent que des emplois stables ne font supporter aucun coût à l'assurance chômage.

toutes les fins de contrats, quelle que soit leur durée, sans distinguer celles qui sont directement imputables à l'entreprise et celles dont elle n'a pas directement la responsabilité. Ainsi, dans la version adoptée à l'Assemblée nationale, une entreprise pourrait être soumise à un malus pour avoir signé des ruptures conventionnelles individuelles ou collectives, alors que ces ruptures nécessitent l'accord du salarié. Ce système n'est pas juste, nous l'avons dit en commission. En refusant l'option de l'à l'américaine, qui était était certes un peu compliquée à mettre en oeuvre, on tombe dans un autre écueil : celui d'un bonus-malus fondé sur le critère trop lâche des fins de contrat. La deuxième raison ignore les paramètres qui seront retenus pour le bonus-malus. Quel sera le périmètre choisi ? Le bonus-malus sera-t-il équilibré uniquement à l'échelon national ou aussi dans chaque secteur d'activité ? Quelle sera l'amplitude de variation de la contribution patronale et sa sensibilité par rapport à la moyenne constatée dans un secteur ? Enfin, la troisième

Quel est le but de l'article 29 sur ce sujet ? Il est de lutter contre la précarité excessive,

Le directeur de l'UNEDIC signale ainsi que « les bénéficiaires de l'assurance chômage qui reprennent des emplois tout en restant inscrits à Pôle emploi présentent des profils variés. Seule une minorité d'entre eux reprend des contrats de moins d'un mois et leur nombre augmente peu. peu. [ ...] « Un diagnostic précis des situations de reprise d'emploi en cours d'indemnisation sera un préalable nécessaire pour étayer les décisions à venir.

de l'effectif total dans les entreprises d'au moins onze salariés, en cas d'accroissement temporaire de l'activité. Le nombre d'embauches en CDD n'a cessé d'augmenter depuis les années quatre-vingt. Ainsi, entre 2000 et 2014, le nombre d'embauches en intérim

que les entreprises connaissent plus souvent des accroissements temporaires d'activité, mais parce que ces contrats sont devenus une variable d'ajustement. De plus en plus de CDD pourvoient durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les exemples ne manquent pas. Ces dernières années, des entreprises comme La Poste ou Air France ont été attaquées à plusieurs reprises par des salariés qui cumulaient des CDD, parfois depuis plus Non seulement le recours excessif aux contrats courts est contraire au droit du travail, qui prévoit que le CDI est la forme normale de la relation de travail, mais il est de plus source de précarité pour les salariés. Les fins de CDD représentent en effet un quart des nouvelles inscriptions à Pôle emploi. Le Gouvernement étend dans le projet de loi les possibilités d'embauche en CDD. Pourtant, M. Macron et sa ministre du travail prétendent vouloir favoriser l'emploi et lutter contre le chômage. Dans cette perspective, ils devraient encadrer strictement les contrats précaires au lieu de faciliter leur utilisation. Afin de lutter contre la précarité et de diminuer les dépenses de l'assurance chômage, nous proposons d'insérer un article additionnel après l'article 29 encadrant le recours aux CDD. Quel

Ce qui mine actuellement les salariés, c'est la précarité, l'instabilité. Aussi, nous proposons ici d'encadrer plus particulièrement le recours aux contrats de travail intérimaires. Il s'agit d'empêcher que ces contrats ne soient utilisés par les entreprises comme un mode de gestion permanent afin que les salariés ne soient pas considérés comme des variables d'ajustement. Nous proposons donc de limiter le nombre de personnes employées en contrat intérimaire à 10 % de l'effectif total dans les entreprises comptant salariés. Certes, cette forme de travail atypique est encadrée par l'article L. 1251-6 du code du travail, mais nous proposons de limiter les possibilités de recours à ce type de contrat aux seuls cas de remplacement d'un salarié absent ou d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Le travail en intérim est augmentation, et ce pour la troisième année consécutive. Au total, 600 000 personnes sont concernées dans notre pays, 600 000 personnes qui n'ont pas de sécurité d'emploi, qui ne savent pas si elles auront encore du travail le mois suivant,

qui ne sont pas vertueuses.

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais. En 2016, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a reconnu pour la première fois la responsabilité sociale des plateformes numériques. Elle impose à ces plateformes de prendre en charge l'assurance couvrant les risques d'accident du travail souscrite volontairement par un travailleur ou un contrat collectif aux garanties équivalentes. Une condition est posée : le travailleur doit avoir réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à 5 100 euros dans l'année, avec une ou plusieurs plateformes. Ce montant est, par exemple, le seuil de déclenchement de l'activité professionnelle pour les locations de meublés ou les tables d'hôtes, en application du décret du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique. Il s'agit donc d'un seuil déjà opérationnel et clairement identifié par les acteurs du secteur. Alors qu'une grève des livreurs des plateformes est en cours, nous vous proposons de créer une allocation spécifique, payée par les plateformes elles-mêmes, contre la perte de revenu pour ces travailleurs, respectant la condition que je viens de mentionner. Cet amendement vise donc à légiférer sur un secteur économique en pleine expansion et qui est appelé à se développer, notamment pour les services à la personne. Il nous apparaît urgent d'élargir le champ de la loi à ces activités boostées par le numérique. Le rapport Terrasse remis en 2016 démontrait bien que l'ubérisation de l'emploi constitue l'un des défis législatifs majeurs de ces prochaines années. Les acteurs du numérique ne peuvent pas continuer à ne suivre que leurs propres lois ou leurs propres chartes ... Mais nous en reparlerons à l'article 40 Dans cette attente, je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement qui constitue une véritable avancée sociale pour ces nouveaux manoeuvriers des temps modernes, qui ne bénéficient à ce jour de presque aucune protection sociale et sont à la merci d'entrepreneurs prédateurs. Les clients ne sont pas en reste et doivent également

Pourtant, notre assemblée se prépare à voter l'article 29 ... En pleine période de chômage de masse, le Gouvernement autoriserait une entreprise à remplacer plusieurs salariés absents

toutefois ensemble les arguments qui ont été développés par le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, et qui nous laissent pour le moins perplexes. Tout d'abord, il s'agirait de couvrir les cas où une seule personne devrait pourvoir à temps plein deux postes vacants à temps partiel. partiel. Les entreprises se retrouveraient alors dans l'impossibilité de recruter. En réalité, ce n'est pas le cas, puisque ladite personne peut tout à fait signer à son tour deux CDD à temps partiel pour occuper les deux postes en question. L'obligation d'un temps minimal de travail de 24 heures hebdomadaires peut par ailleurs être contournée sur seule déclaration du salarié en cause. Il s'agirait ensuite de permettre le remplacement de deux personnes employées successivement, en couvrant par un seul contrat les deux périodes concernées. Mais, une nouvelle fois, la situation actuelle est tout à fait vivable, puisque la succession de CDD est aujourd'hui monnaie courante. Au final, la seule justification à cet article est une nouvelle fois de précariser la situation des salariés en CDD et de limiter les coûts pour les entreprises. En effet, la rédaction de l'article, même après sa transformation par la commission des affaires sociales, est tellement large que toute entreprise pourrait remplacer dans tous les cas plusieurs salariés.

Ensuite, elle sera limitée à des secteurs définis par un décret qui devrait être pris avant le 1 janvier 2019. En outre, la durée de l'expérimentation sera réduite à deux ans avant une éventuelle généralisation. Par ailleurs, afin d'éviter tout risque de contournement des règles d'ordre public social en matière de contrats courts, les CDD et contrats d'intérim multi-remplacements ne pourront pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale ou permanente de l'entreprise. Enfin, l'évaluation de l'expérimentation devra se pencher sur les nouvelles compétences reconnues aux partenaires sociaux de branche depuis l'ordonnance Travail du 22 septembre 2017.

Lavarde. Le recours aux contrats d'usage dits « extras » est une nécessité, par exemple dans la branche de l'hôtellerie et de la restauration, afin de faire face aux fluctuations d'activité. Une jurisprudence de la Cour de cassation de septembre 2008 considère que la seule qualification conventionnelle de « contrat d'extra » impose de rechercher, pour l'emploi considéré, non seulement s'il est effectivement d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mais également si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives. Or la preuve du caractère par nature temporaire de l'emploi est en réalité impossible à fournir. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main-d'oeuvre résultant d'un événement particulier, par exemple une réception En revanche, les métiers qui sont confiés à ces salariés employés en extras- serveurs, maîtres d'hôtel -ne sont évidemment pas temporaires par nature. Aussi, faute de pouvoir apporter la preuve du caractère par nature temporaire de l'emploi, et même si l'employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient le CDD en le CDD en CDI et la relation de travail à temps partiel en temps complet. Ces décisions aboutissent à des condamnations de plusieurs centaines de milliers d'euros. Cet amendement, s'il était adopté, permettrait donc de définir dans le code du travail la notion d'emploi par nature temporaire dans les secteurs d'activité définis par décret ou accord de branche.

l'avis du Gouvernement ? Il est défavorable. Cet amendement vise à modifier les textes qui définissent les cas de recours aux CDD d'usage, notamment pour « contrecarrer » une jurisprudence de la Cour de cassation sur l'utilisation de ce type de contrats dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Je vous l'accorde, la réglementation sur le CDD d'usage est un peu complexe, car elle se situe au confluent des réglementations française et européenne, notamment avec la directive concernant les CDD.

En outre, et c'est peut-être le point le plus important, la réforme récente a ouvert à la négociation des partenaires sociaux la question du calcul et de la suppression du délai de carence, ce qui est de nature à répondre à cette problématique.

Avec cet amendement, nous vous proposons de renforcer les droits des salariés au sein des comités d'entreprise encore en place dans certaines entreprises et dans les nouveaux comités sociaux et économiques, les CSE, créés par les ordonnances dites « dialogue social ». Je rencontre

: ce serait bien que, à la fin de l'année, on puisse faire le bilan de la mise en place des CSE, car de nombreux syndicalistes sont inquiets. Nous pensons que les représentantes et représentants des salariés doivent être consultés chaque année pour donner un avis conforme sur le recours aux entreprises de travail temporaire et aux contrats de travail à durée déterminée. Désormais, les comités d'entreprise et les comités sociaux et économiques pourront formuler des propositions complémentaires ou alternatives au projet de l'employeur.

des études et des statistiques, la part des embauches en CDD a fortement progressé en vingt-cinq ans, passant de 76 % en 1993 à 87 % l'an dernier, et que, entre 2001 et 2017, la durée moyenne d'un CDD en France a été divisée par plus de deux, passant de 112 jours à 46 jours. L'avis conforme du comité d'entreprise sur le recours aux formes précaires de contrats de travail permettrait de prévenir de manière efficace le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail, ce qui paraît d'autant plus nécessaire qu'un tiers des CDD ne dure qu'une seule journée. Afin de prévenir de manière effective le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail, nous estimons que rendre obligatoire pour les employeurs l'avis conforme du comité social et économique serait une solution aux problèmes que nous rencontrons. Quel

perturbent la discussion de cet article 30. La suppression des contributions chômage salariales et leur remplacement par l'augmentation du taux de la contribution sociale généralisée, la CSG, sociale pour 2018 entraînent une bascule du financement de la sécurité sociale par les cotisations vers l'impôt, ce qui est contraire à l'esprit de la sécurité sociale. Avec cette réforme, l'État prend désormais en charge 45 % du total des ressources de l'assurance chômage, si l'on ajoute les 13,6 milliards d'euros de contribution chômage des salariés et les 3 milliards d'euros de contribution chômage des employeurs, anciennement pris en charge par le CICE, L'étatisation de l'assurance chômage est, selon nous, un danger, car elle va entraîner la disparition du paritarisme de la sécurité sociale, qui est pourtant l'un des fondements de notre système avec une gestion en commun des organismes sociaux par les représentants des salariés et ceux du patronat, du financement contributif à l'assurance chômage par le biais de cotisations salariales et patronales assises sur les salaires, élément fondamental de notre système d'assurance sociale, et, enfin, de notre système assurantiel, qui va basculer vers un système d'assistance dans lequel les prestations seront remplacées par des droits auxquels s'ajouteront des devoirs.

au titre de la majoration spécifique. Cette majoration de la part des contributions chômage à la charge des employeurs a été mise en place pour les CDD d'usage inférieurs à trois mois et a été prorogée, en octobre 2017, jusqu'au 31 mars 2019. Dès lors, il nous semble inéquitable de soumettre ces contrats à la possibilité d'une modulation supplémentaire, qui serait fondée sur un même critère. C'est pourquoi notre amendement vise à exclure ces contrats de la modulation résultant de l'application du 2° de l'article L. 5422-12 du code du travail.

Laurence Cohen, sur l'article. La suppression des cotisations salariales et les exonérations de cotisations patronales ont entraîné une augmentation de la participation de l'État aux recettes de l'assurance chômage qui est désormais de de plus de 40 %. L'État veut par conséquent participer aux négociations de l'UNEDIC à la hauteur de sa participation financière. L'article 32 prévoit donc le renforcement du rôle de l'État, puisque le Premier ministre fixera avant les négociations collectives, la trajectoire financière du régime d'assurance chômage, le délai dans lequel ces négociations doivent aboutir et les objectifs d'évolution des règles de ce régime. Et si les résultats de la négociation sociale ne respectent pas ce document, le Gouvernement pourra fixer directement les règles de l'assurance chômage par décret. Cette reprise en main par l'État du pilotage du régime d'assurance chômage

paroles ! Dans ce cadre, les partenaires sociaux n'auront plus qu'un rôle subalterne : appliquer sans marges de manoeuvre financières la feuille de route dictée par un gouvernement qui vante pourtant les mérites du dialogue social. On soumet ainsi l'assurance chômage à une logique comptable, de la même manière que l'on gère le budget de l'assurance maladie sans tenir compte déplorons. Sans possibilité d'agir sur le volet « recettes », il est à craindre que les partenaires sociaux ne soient enfermés dans un cercle vicieux, qui les amènera à réduire les dépenses, donc l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. Pour conclure, les attaques contre notre sécurité sociale ne cessent de pleuvoir durant ce quinquennat, comme l'illustre l'amendement d'un député du groupe La République En Marche visant à retirer la référence à la sécurité sociale dans la Constitution.

Savoldelli. Depuis 1958, les organisations représentatives des salariés et des employeurs cogèrent le système de protection contre la privation involontaire d'emploi- La loi garantit le bon fonctionnement et le financement du régime d'assurance chômage. Concrètement aujourd'hui, les syndicats de salariés et les employeurs négocient ensemble pour déterminer les objectifs et les principes de l'assurance chômage pour une durée limitée de deux ou trois ans. Le document qui en découle, la convention d'assurance chômage, est soumis ensuite à l'agrément du ministère chargé de l'emploi, afin de vérifier sa conformité avec les normes juridiques et les actions menées en matière d'emploi. Enfin, l'agrément ministériel rend obligatoire la convention, qui s'applique directement aux salariés et aux employeurs. Demain, avec cet article 32, le Premier ministre devra transmettre un document de cadrage

Et si les résultats de la négociation sociale ne respectent pas ce document ou si la situation financière se détériore en cours d'année, le Premier ministre pourra retirer l'agrément de l'accord portant convention d'assurance chômage et prendre lui-même les mesures d'application du régime d'assurance chômage. L'encadrement par l'État des négociations sociales de l'assurance chômage ne laisse presque plus de place aux syndicats et au patronat.

C'est une différence essentielle en termes de logique et de responsabilité.

qu'il ne s'agit là que d'une faculté, le document de cadrage pouvant très bien se limiter à fixer un objectif pour la trajectoire financière, sans intégrer ce deuxième volet. Quel est l'avis

de loi qui instaure l'expérimentation d'un journal de bord, dans lequel les demandeurs d'emploi devront rendre compte mensuellement de leurs actions de recherche à l'occasion du nouvellement de leur demande d'allocation. Une telle expérimentation vise à accroître le contrôle des demandeurs d'emploi, pourtant déjà très fort.

Renforcer le contrôle des chômeurs présente plusieurs conséquences négatives. D'abord, cela contribue à transformer les conseillers de Pôle emploi en agents de contrôle. Un tel contrôle demande un investissement temporel démesuré au regard du faible taux de fraude. De plus, le rôle des conseillers de Pôle emploi consiste à accompagner les demandeurs d'emploi, pas à constater mensuellement l'échec des actions de recherche Pointer du doigt les chômeurs et renforcer les contrôles à leur égard nous font oublier que le chômage est un droit, pas un cadeau accordé par l'État. Chaque mois, plutôt que de recevoir la totalité de leur salaire, les salariés en consacrent une partie au financement de l'assurance chômage. Cette démarche Cette démarche leur permet de bénéficier d'un salaire différé, disponible dans l'éventualité où ils perdraient leur emploi. Le droit à l'allocation chômage dépend donc des cotisations, et pas des efforts fournis par les demandeurs d'emploi pour retrouver un travail. Ceux qui bénéficient du chômage de plein droit ne devraient par conséquent pas avoir à prouver leurs actions de recherche. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Je suis défavorable à cet amendement, parce qu'un amendement relatif à la remise d'une évaluation de l'expérimentation du journal de bord a déjà été adopté en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. De plus, le délai proposé dans le présent amendement est postérieur au terme de l'expérimentation. Il suffit de revenir au texte initial et tout est résolu.

et les chiffres le prouvent. Pour 2016, Pôle emploi a ainsi évalué le nombre d'emplois vacants, c'est-à-dire des recrutements abandonnés faute de candidats correspondant au poste, entre 200 000 et 330 000. 330 000. Au quotidien, nous avons tous des exemples de postes non pourvus dans nos départements : soudeurs, chaudronniers, plombiers, notamment, des métiers qui recrutent, aux salaires intéressants, mais qui souffrent d'une mauvaise image, L'amendement que nous présentons vise à donner un nouveau souffle à un dispositif utile face à cette situation, mais assez peu utilisé : la mise en situation en milieu professionnel. Ce dispositif permet des immersions de courte durée et de découverte. Quoi de mieux que vivre le métier au quotidien pour apprécier ses valeurs, son univers, pour le comprendre et savoir s'il nous convient ? Ce dispositif devrait être axé non seulement sur les métiers en tension, mais aussi sur les métiers d'avenir, qui recruteront le plus, par exemple, les métiers de l'intelligence artificielle. Nous pensons, par ailleurs, que les branches professionnelles devraient oeuvrer à une meilleure connaissance de ce dispositif d'immersion,

Le Gouvernement soutient leur développement, en particulier dans les métiers en tension, mais pas que. Il ne faut pas être restrictif sur le sujet.

Cet amendement vise à réécrire l'article 35, afin, d'une part, de supprimer les dispositions qu'il introduit, et, d'autre part, d'abroger l'article L. L. 5411-6-2 du code du travail, qui définit la notion d'offre raisonnable d'emploi. Lors du premier entretien à Pôle emploi, un demandeur d'emploi et son conseiller vont définir l'offre raisonnable d'emploi. Les critères de cet emploi, tels que la nature et les caractéristiques de celui-ci, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu sont alors précisés. raisonnable d'emploi type sera différente selon les candidats et les profils. Sa détermination est censée permettre au demandeur d'emploi d'exprimer ses souhaits concernant l'emploi recherché. En réalité, ce dispositif permet un contrôle accru du demandeur d'emploi. En effet, le présent projet de loi prévoit que celui-ci n'a le droit de refuser qu'une fois un emploi qui entrerait dans le cadre de son offre raisonnable. Au-delà, il pourra être radié du chômage, c'est-à-dire qu'il pourra perdre ses indemnités et se retrouver sans ressources. Autrement dit, l'offre raisonnable d'emploi permet de contraindre les demandeurs d'emploi à accepter des offres qui ne leur conviendraient pas, sous la menace d'une sanction. Il est important de rappeler que l'allocation chômage constitue un salaire différé. Chaque mois, les salariés, plutôt que de toucher l'intégralité de leur salaire, en consacrent une partie au financement de l'assurance chômage, sous forme de cotisations sociales. Les indemnités versées par l'assurance chômage sont donc non pas un cadeau de l'État accordé aux chômeurs, mais tout simplement du salaire épargné par les salariés. Les demandeurs d'emploi devraient pouvoir disposer librement de leur salaire différé, sans avoir à justifier de leurs agissements.

des sanctions éventuelles à l'égard d'un demandeur d'emploi de la situation du marché local. Cela voudrait dire que, selon l'endroit où l'on habite,

L'avis de la commission 35 vise bien une information du demandeur d'emploi à l'occasion de la mise en place du PPAE, ce qui nous semble nécessaire, notamment parce que nous sommes en période de croissance.

à l'emploi se négocie avec Pôle emploi, et il définit les conditions dans lesquelles l'emploi doit être accepté, l'intéressé

vous avez une connaissance parfaite du sujet- je suis admiratif -, mais vous avez aussi parfois une vision un peu angélique de la relation qui peut s'établir entre le demandeur d'emploi et Pôle emploi. Il ne faut pas oublier que pèse toujours la

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Cet article durcit les cas de suspension de l'allocation chômage. Par exemple, la simple absence du demandeur d'emploi à un rendez-vous ou à une formation pourra être sanctionnée, sans qu'il soit précisé s'il peut justifier son absence ou si certains motifs sont acceptables, un problème de santé par exemple. Actuellement le demandeur d'emploi ne peut être sanctionné qu'en cas de refus de se présenter. Cet article durcit également le contrôle des chômeurs, puisqu'un renforcement de l'accompagnement du demandeur d'emploi peut être décidé lorsque ce dernier a fait l'objet d'une radiation. Celle-ci pourra d'ailleurs durer entre un et six mois en cas de manquement ; elle pourra même être définitive. Enfin, les sanctions pécuniaires sont renforcées, puisque leur montant maximal passe de 3 000 à 10 000 euros. L'application de ces nouvelles sanctions va nécessairement entraîner un surcroît d'activité pour les conseillers de Pôle emploi, alors même que ce projet de loi prévoit une diminution du personnel et une baisse des moyens. À ce sujet, il paraît important de rappeler que la fraude à Pôle emploi représente seulement 0,5 % des allocations versées, selon un rapport de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude. Il est certain que le temps et l'argent investis dans cette

C'est d'ailleurs le seul et unique rôle que les conseillers de Pôle emploi devraient assumer, puisque l'allocation chômage est non pas une faveur que l'État accorde au demandeur d'emploi, mais bien un droit tiré des cotisations sociales. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression partielle de l'article 36. L'amendement

Le scrutin est ouvert.

La chambre sociale de la Cour de cassation a retenu la caractérisation de la négligence fautive de l'organisme chargé de verser des allocations d'assurance chômage. Lorsque

il me semble que cet amendement n'est pas justifié, du fait, précisément, que le principe de la responsabilité civile est d'ordre législatif et d'application générale. L'article 1240 du code civil

des complexités administratives qui peuvent décourager les demandeurs, ou tout simplement la honte. Je vous rappelle que le Défenseur des droits lui-même s'est inquiété de ces non-recours qui placent des personnes déjà précaires dans des situations encore plus délicates. Il s'agit d'un phénomène de société complètement sous-estimé, et je pense, tout comme mon groupe, que ces non-recours ont aussi un coût au final et qu'il serait donc utile de les limiter et d'inciter davantage les bénéficiaires potentiels à effectuer les démarches. Notre amendement, circonscrit aux droits en matière d'assurance chômage, vise, par exemple, un défaut d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi ou bien de recours aux droits par les demandeurs d'emploi. Quel est l'avis

Cathy Apourceau-Poly. En cohérence avec notre amendement de suppression de l'article 32, nous proposons la suppression de l'article 37. En effet, nous ne pouvons accepter cette remise en cause du caractère paritaire de l'UNEDIC et le retrait de l'intervention des partenaires sociaux dans la gestion de l'assurance chômage. L'article 37 se résumant à la mise en oeuvre de cette réforme dans les outre-mer, il est donc normal que nous demandions sa suppression. Quel

nécessaires à la vérification de la validité des titres de séjour et de travail des personnes étrangères lors de leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Cette inscription a plusieurs effets : elle exonère l'employeur embauchant un étranger inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de la vérification de l'existence du titre autorisant l'intéressé à exercer une activité salariée en France. Par le biais de cet amendement, nous proposons que la transmission d'informations puisse avoir lieu en cas de renouvellement des titres de séjour et de travail qui ont

L'intermédiation numérique comme activité spécifique justifierait une telle mise à l'écart : il n'y aurait plus de travailleurs et encore moins de salariés, mais des utilisateurs ou des prestataires extérieurs ; il n'y aurait plus d'employeurs, mais des intermédiaires, plus de sanctions directes, mais des incitations et la désactivation fait figure de rupture contractuelle « euphémisée ». Il ne s'agit pourtant que d'une torsion de la réalité opérée par le recours à un langage spécifique. Dans les faits se multiplient les pratiques de concurrence déloyale envers les entreprises qui respectent la loi et s'observe une vaste opération de dumping social. La Cour de justice de l'Union européenne est pourtant formelle : l'intermédiation numérique n'est que la modalité d'exécution d'un service qui dépasse la simple mise en relation. Si Uber est une société de transport, Deliveroo une société de livraison de repas, ces plateformes ont besoin de travailleuses et de travailleurs qui réaliseront pour leur compte l'activité économique et commerciale qu'elles encadrent et dirigent. C'est ce qu'on appelle du travail salarié. Or le développement des plateformes numériques de travail est l'occasion d'une paupérisation terrible des travailleuses et des travailleurs, à l'écart du statut de l'emploi, payés à la tâche, sans assurance maternité, chômage, vieillesse ou maladie, sans protection contre le pouvoir de contrôle, de direction et de sanction des plateformes, soumis à la loi du plus fort. Pour protéger ces travailleurs, lutter contre le faux travail indépendant, le dumping social et les pratiques de concurrence déloyale, il semble alors indispensable d'établir une présomption de salariat qui explicite la nature de l'état de subordination, ainsi que de mieux identifier le débiteur des obligations légales et contractuelles par une définition de l'employeur. L'amendement Le développement des technologies numériques a d'ores et déjà modifié en profondeur les organisation et mode de travail de très nombreux actifs. L'essor de ce que l'on appelle désormais le travail à la demande, que traduit l'avènement des plateformes numériques, a indéniablement contribué à l'accélération de cette évolution. Les plateformes collaboratives présentent néanmoins une ambivalence : d'un côté, elles offrent des opportunités d'activité pour de nombreux actifs, qu'il convient d'accompagner de l'autre, leur modèle de fonctionnement fragilise ces mêmes actifs, qui, s'ils sont officiellement non subordonnés à la plateforme, restent néanmoins dépendants économiquement. Les fortes perspectives de développement de ce secteur et la fréquence des conflits sociaux en son sein appellent une réaction. Depuis le début de la semaine, des livreurs de plusieurs plateformes de livraison de repas sont en grève pour protester contre la précarisation de leur statut. La multiplication, La multiplication, ces derniers mois, de tels mouvements des travailleurs de plateformes doit être perçue comme une alerte qui nous est adressée. Mes chers collègues, il incombe aux responsables politiques de prendre acte des changements profonds qu'opère la révolution numérique au sein de notre société et d'accompagner ces derniers. La sécurisation de la relation entre les plateformes et les travailleurs indépendants et le développement de la responsabilité de ces plateformes doivent être une Dans ce contexte, vous l'aurez bien compris, l'établissement d'une charte des plateformes destinée à rendre effective cette responsabilité et à protéger davantage les travailleurs indépendants paraît indispensable.

Il revient en effet à la puissance publique de fixer le statut de ces travailleurs et d'assurer ainsi leur protection. Or voilà que le groupe La République En Marche entend réintroduire ce dispositif. Nous ne sommes pas dupes : c'est bien parce qu'une célèbre plateforme de livraison de repas risque de voir requalifier en relation salariée le contrat de certains de ses livreurs que ce « cavalier » arrive en discussion. vise à une protection, c'est bien à celle des plateformes et non à celle de leurs travailleurs. Mais les travailleurs de l'ubérisation de notre société doivent, comme tous les autres, relever du code du travail. D'ailleurs, un mouvement en ce sens a été engagé, notamment avec la protection contre les accidents du travail et le droit à la formation qui leur ont été reconnus dans un chapitre spécifique du code du travail relatif à la responsabilisation sociale des plateformes. Actuellement, des livreurs parisiens de ces plateformes sont en grève pour obtenir de meilleures conditions de travail, car, à ce stade, ils représentent le sous-prolétariat du XXI siècle. En nous opposant à cet amendement, nous nous faisons le relais de ces tâcherons modernes, comme ils se définissent eux-mêmes, qui jugent que votre démarche va renforcer l'arbitraire du secteur et pérenniser la précarité. D'ailleurs, ils ont directement interpellé le parlementaire à l'initiative de cet amendement, le député Aurélien Taché, qui n'a pas jugé utile de les recevoir afin d'entendre leur point de vue. La parole est à M.

La sous-traitance en cascade est un fléau pour la santé économique de nos entreprises et pour le principe de justice sociale qui devrait guider les actions politiques. Alors que la sous-traitance ne devrait être que le moyen de confier la réalisation d'un ouvrage à des personnes disposant de compétences particulières et d'un savoir-faire spécifique, elle s'est révélée être un redoutable outil de fragmentation de l'entreprise, l'expression de stratégies d'externalisation productive à des fins de coût. La multiplication des niveaux de sous-traitance est en effet un moyen pour faire des économies. À chaque niveau, une entreprise donneuse d'ordres fait ainsi pression sur son sous-traitant pour maximiser ses marges et limiter ses risques, en les faisant porter sur d'autres. En bout de chaîne, les petites entreprises et les artisans sont asphyxiés et contraints à réduire la qualité des produits et, surtout, à faire travailler les salariés dans des conditions dégradées. Sur un même lieu de travail se multiplient ainsi les statuts salariaux. Pour une même activité, les salaires, les garanties contractuelles individuelles ou le niveau des protections collectives varient, provoquant d'injustes et d'inexcusables inégalités de traitement. L'Allemagne et l'Espagne, pour ne prendre que ces exemples européens, ont légiféré bien avant nous sur la limitation Cette limitation permet non seulement aux droits des travailleurs d'être mieux identifiés et mieux respectés, mais aussi de restreindre les situations de dumping social, de concurrence déloyale, et ainsi d'agir pour la santé de notre tissu économique, la stabilité de l'ordre public et l'impératif de justice sociale. Cet amendement s'inscrit dans cette dynamique d'identification et de sécurisation, à la fois des salariés, mais également des entreprises sous-traitantes. Les limites du modèle taylorien du travail ont largement été atteintes avec ce développement de la sous-traitance. Aussi, il est proposé d'encadrer cette pratique en la limitant à deux échelons et de la soumettre aux instances représentatives du personnel, chargées de déterminer s'il s'agit d'une opération d'externalisation ou si les compétences attendues sont bien absentes de l'entreprise donneuse d'ordres. Quel est l'avis de la commission

du chapitre du projet de loi qui s'attache à rendre les entreprises plus inclusives, je souhaite rappeler quelques chiffres importants : 2,7 millions de personnes en âge de travailler sont en situation de handicap, mais trente ans après la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le taux d'emploi direct dans les entreprises du secteur privé est de 3,4 % pour un objectif de 6 %. Il atteint 5,2 % dans la fonction publique. Par ailleurs, le chômage des travailleurs handicapés reste trop élevé, avec un taux de 19 %. Face à ces constats, la mobilisation globale de l'État, des partenaires sociaux, des associations et des entreprises doit être maximale pour refuser ce qui après trente ans pourrait s'apparenter à de la résignation, voire à de la fatalité. Aussi, je tiens à saluer le travail de concertation conduit par vous-même, madame la ministre, et par Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, ainsi que le précieux travail par Dominique Gillot sur l'emploi des travailleurs handicapés et sur les aidants qui va continuer de nourrir la deuxième phase de concertation jusqu'au mois de septembre. Je veux également souligner l'importance pour mon groupe de réintroduire l'entreprise comme périmètre de calcul de l'obligation d'emploi, sans autre condition de seuil. Il s'agit pour nous d'une disposition importante et le seuil de 250 salariés adopté par la commission n'est pas acceptable à nos yeux. Il priverait la nouvelle échelle de calcul de l'essentiel de son effet, alors que, je le répète, la mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés doit

Il existe également un frein psychologique à l'emploi. En effet, les entreprises considèrent trop les personnes handicapées du point de vue de leur handicap, de leur limitation, plutôt que du point de vue de leurs compétences. L'article 40 et les suivants du projet de loi prévoient de réformer la politique de l'emploi en faveur des travailleurs handicapés. Mais sommes-nous réellement devant une vraie réforme ou face à un coup de communication ? En effet, ? En effet, de nombreuses mesures proposées ressemblent fort à l'état du droit actuel et s'apparentent bien souvent à des allégements pour les entreprises, notamment concernant l'acquittement de l'obligation d'emploi, peu favorable à l'emploi direct. Comme sur beaucoup d'autres textes de loi présentés par le Gouvernement, des négociations parallèles sont toujours en cours et, parfois, aboutissent. Hier, une convention très engageante a été signée en vue de doubler d'ici à 2022 le nombre de créations d'emplois dans le secteur adapté. Mais, en même temps, si j'ose dire, le Gouvernement réduit drastiquement la prime d'activité pour les salariés percevant une pension d'invalidité ou une rente accident du Cette mesure d'économie de 20 millions d'euros plonge des centaines de familles, notamment monoparentales, dans la misère. D'un côté, le Gouvernement nous annonce des lendemains qui chantent à l'horizon de la fin du quinquennat. Et, de l'autre, il coupe les vivres aux personnes en situation de handicap les plus fragiles et les plus modestes ! Quelle contradiction Je ne vois pas en quoi les mesures proposées dans le présent projet de loi sont de nature à contrebalancer la suppression indigne de la prime d'activité pour les personnes handicapées les plus faibles. Enfin, des inconnues de taille demeurent sur les questions relatives à la contribution, à son montant ou barème et à ses modalités de recouvrement par l'URSSAF. Il manque véritablement une étude d'impact.

par tous les employeurs. Le rapport de Dominique Gillot insiste, lui aussi, sur la nécessité de prendre en compte le maintien en emploi comme un moyen pour lutter contre la désinsertion professionnelle et comme un levier essentiel pour favoriser la sensibilisation des employeurs. C'est pourquoi nous vous proposons d'ajouter cette mention. Au-delà de la mobilisation pour l'emploi dans le cadre de la généralisation de la déclaration sociale nominative, la fameuse DSN, à tous les employeurs, celle-ci doit s'inscrire dans une démarche pérenne d'ouverture à l'égard de l'emploi des personnes en situation de handicap. Quel

En revanche, son objet soulève un point intéressant : faire apparaître dans la DSN l'objectif de maintien dans l'emploi des personnes handicapées, par opposition avec l'embauche stricte.

toutes les capacités, toutes les compétences des personnes handicapées et leur volonté d'accéder au travail. C'est un changement de paradigme parce que, de manière positive, nous voulons inciter les entreprises à prendre en considération toutes les palettes que nous leur offrons avec cette rénovation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

amendement. La précision selon laquelle la mobilisation des employeurs concerne également le maintien en emploi des travailleurs handicapés n'est pas nécessaire puisque l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés recouvre par essence même à la fois le recrutement des personnes handicapées et le maintien